L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée,

L'argument principal avancé en faveur de la création de ce fichier d'enfants, car c'est bien de cela qu'il s'agit, est le suivant : « Les coûts imposés aux départements lors de la phase d'évaluation de la minorité sont très supérieurs à la compensation accordée par l'État ». En résumé, l'argument est donc financier ... Il est vrai que, au titre de leurs compétences en matière de protection de l'enfance, les départements sont en première ligne : ils ont en effet réalisé plus de 54 000 évaluations sociales préalables à la confirmation de la minorité. Toutefois, la mise en oeuvre du mécanisme d'évaluation de l'âge et de l'isolement de ces jeunes s'est transformée en une opération pour séparer le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire débusquer les jeunes majeurs- prétendument majoritaires -des véritables mineurs. Or tous ces jeunes sont en situation de détresse Sans parler des méthodes contestables de reconnaissance, qui passe souvent par des tests osseux ou des entretiens réalisés dans de très mauvaises conditions, la création d'un tel fichier déshonore notre pays, en marquant au fer rouge des exilés qui, s'ils ne sont pas effectivement mineurs, sont dans la plupart des cas de très jeunes adultes vulnérables qui ont connu un parcours migratoire terrible et viennent chercher refuge dans notre pays. Aucune de ces personnes vulnérables, mineure ou majeure, ne mérite d'être ainsi fichée. C'est pourquoi nous sommes absolument opposés à la création d'un nouveau fichier, pour des enfants. Au regard de la nature des données visées, des risques de détournement de ces données et de l'usage illicite qui pourrait en être fait, nous pensons qu'un tel outil porte nécessairement une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, ainsi qu'à la protection des données personnelles. La création de ce fichier fera courir le risque d'une exploitation étrangère à l'objectif affiché, à savoir

à la problématique des mineurs non accompagnés, dont le rapporteur vient de rappeler la double importance : d'une

accord : tout en maintenant la compétence des départements dans l'évaluation et la prise en charge des mineurs, l'État peut leur apporter une contribution plus déterminante en ce qui concerne l'évaluation préalable de la minorité. Parmi les solutions proposées Parmi les solutions proposées et arrêtées figure la création d'un traitement automatisé de données, afin de contribuer à l'identification des personnes étrangères se disant mineurs non accompagnés, de mieux garantir la protection de l'enfance et d'éviter que des personnes reconnues majeures ne fassent l'objet d'évaluations successives de minorité dans d'autres départements, comme le rapporteur À la demande des présidents de conseil départemental, les demandeurs seraient reçus en préfecture par des agents ayant la charge de renseigner ce fichier. Sa création s'accompagnerait d'importantes garanties de respect de la vie privée, avec notamment une courte durée de conservation des données.

Or il convient de promouvoir la collecte des données de tous les demandeurs, et non celles des seuls majeurs, pour toute la durée de l'évaluation, afin de pouvoir procéder à leur identification à un stade précoce et d'éviter la multiplication postérieure En outre, la création d'un traitement automatisé de données personnelles est régie par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui prévoit qu'un tel traitement est créé par la tel traitement est créé par la voie réglementaire après, le cas échéant, un avis de la CNIL. Il importe que la procédure soit respectée afin que soit pleinement appréciée la proportionnalité du traitement envisagé au regard, notamment, des finalités recherchées et de la nature des données.

concerne le droit d'asile, l'immigration et l'intégration des étrangers, il n'y a pas lieu d'y introduire des dispositions qui relèvent d'autres législations, par exemple le code de l'action sociale et des familles. C'est pourquoi le Gouvernement estime, sur

Pour l'ensemble des raisons qui ont été très bien expliquées précédemment, y compris, d'ailleurs, par Mme la ministre, mais aussi évidemment par les auteurs des amendements identiques, nous voterons en faveur de la suppression de cet article.

observer les conditions dans lesquelles ces supposés mineurs, qui ne le sont pas toujours, arrivent dans nos départements. Vous avez raison de le souligner dans l'objet de l'amendement, ces jeunes ont eu un parcours extraordinairement difficile, c'est vrai,

! ... équipés de pieds en cap de maillots de football, de baskets, de téléphones, fournis non pas par les services départementaux, mais par les passeurs eux-mêmes. C'est ce qui nous a été rapporté dans les Hautes-Alpes et nous sommes six sénateurs à avoir entendu la même chose. Il suffit d'un minimum d'objectivité et de courage,

Il n'est tout de même pas acceptable que les départements ne puissent pas avoir accès à un fichier qui leur permette de savoir si, éventuellement, la personne qui se présente devant eux

est en discussion, laissons faire les choses, occupons-nous de ce qui nous regarde. En la matière, le Sénat ferait oeuvre de bonne législation en adoptant ce principe. Je

la fiabilité scientifique des tests osseux pratiqués sur les jeunes étrangers destinés à déterminer leur âge est aujourd'hui contestée. Dans ces conditions, il est proposé de ne pas verser le résultat de ces tests dans le traitement automatisé de données créé par l'article 26

n'est qu'un élément parmi d'autres.

Or, le contrat jeune majeur étant un dispositif sur lequel le département exerce une compétence discrétionnaire, son attribution à un jeune majeur anciennement mineur non accompagné n'a d'autres motifs que la volonté d'intégration que montre l'attributaire et le désir du département d'«investir » pour sa réussite. Il s'agit donc d'une démarche qui, en raison de son caractère subsidiaire, suffit à prouver la confiance portée par les pouvoirs publics au demandeur du titre. Par ailleurs, à l'heure actuelle, en refusant l'admission au séjour à un titulaire d'un contrat jeune majeur sur ce seul motif, l'autorité préfectorale annihile tout bonnement les efforts déployés par le département en vue de l'intégration de ce jeune. En plus d'interrompre le parcours d'intégration, le refus d'admission représente pour les départements un aléa important, susceptible de freiner l'attribution de ces contrats à d'anciens mineurs non Par conséquent, il semblerait judicieux que l'admission d'un jeune majeur isolé à un dispositif de protection sociale subsidiaire financé par le conseil départemental puisse être favorablement considérée à l'appui de sa demande d'admission au séjour.

Si les jeunes accueillis avant seize ans peuvent être considérés comme une catégorie relativement homogène- ils comptent deux ans au minimum de présence en France avec un accompagnement par les services du département

très peu accompagné. L'assouplissement des conditions d'admission au séjour n'est donc pas souhaitable dans le contexte actuel de recrudescence d'arrivées importantes de mineurs non accompagnés sur le territoire français. Ouvrir à tous ceux qui sont accompagnés par l'ASE, y compris depuis quelques semaines seulement, l'admission au séjour, de surcroît sans examiner la situation de manière globale et sans tenir compte des liens conservés avec la famille restée dans le pays d'origine, pourrait conduire à régulariser un jeune majeur

avec la famille restée dans le pays d'origine pour les étrangers confiés à l'ASE entre seize et dix-huit ans et entrant dans le champ d'application de l'article L. 313-15 du CESEDA. En effet, une circulaire du ministère de l'intérieur ministère de l'intérieur indique que l'autorité administrative n'a pas à opposer systématiquement le critère tiré de la nature des liens avec le pays d'origine. Toutefois, on constate que les préfectures ont des pratiques très diverses et que certaines d'entre elles

L'amendement n° 362 rectifié vise à protéger plus spécifiquement les mineurs, en complétant le protocole organisant une réponse globale en matières éducative, culturelle et sociale, de santé et de logement.

avait estimé ces dispositions contraires au droit au recours juridictionnel effectif, puisqu'aucune règle générale de droit français ne prévoit de recours contre les décisions du parquet devant une juridiction. La commission comprend l'intention des auteurs de cet amendement, qui s'interrogent sur la capacité des autorités françaises de procéder à la réadmission dans

Il est impossible de déjudiciariser le renvoi des enfants mineurs dans leur pays. La protection de l'enfant est une obligation de l'État constitutionnellement garantie. C'est toujours le juge des enfants, par ordonnance judiciaire,

afin « d'en aménager le plan, d'en clarifier la rédaction et d'y inclure les dispositions d'autres codes ou non codifiées relevant du domaine de la loi et intéressant directement l'entrée et le séjour des étrangers en France Après le code du travail, après la réforme du secteur ferroviaire, il s'agit donc ici de récrire le code consacré à la politique migratoire et d'asile par voie d'ordonnance. Nous sommes opposés à une telle habilitation. Ce sujet mérite un examen précis par le Parlement. Une nouvelle codification, même si ses motifs sont purement formels, n'est jamais anecdotique : elle emporte toujours de l'implicite, sur lequel le Parlement devrait pouvoir statuer sereinement, sans donner mandat au Gouvernement. Cet article vise également à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour simplifier le régime des autorisations de travail pour le recrutement de certaines catégories de salariés par des entreprises bénéficiant d'une reconnaissance particulière de l'État.

Cet amendement vise à rétablir les habilitations à modifier le CESEDA par ordonnance qui ont été supprimées par la commission des lois

». La coexistence de ces deux cartes de séjour intéressant des publics aux caractéristiques proches est à l'origine d'une grande complexité. Éclairé par des échanges réguliers avec les professionnels et les partenaires sociaux, particulièrement demandeurs de cette modification, le Gouvernement souhaite simplifier le régime de ces deux cartes de séjour en les fusionnant. La mise en place de ce nouveau régime réclamera un certain délai, notamment du fait de la consultation de plusieurs organismes publics et privés- Pôle emploi, par exemple -, afin de mettre en place un mécanisme complet et adapté aux besoins du marché, des employeurs et des salariés.

Là encore, le Gouvernement souhaite pouvoir revoir le régime des autorisations de travail dans toutes ses dimensions : objectif, conditions de délivrance, procédure, contrôles. Un groupe de travail interministériel a d'ailleurs été créé sous l'égide du ministère de l'intérieur pour avancer sur cette thématique. Ses travaux permettront de définir un dispositif juridique complet et opérationnel adapté au nouveau contexte économique et du marché du travail. Quel

dans la vie politique, en atteste. En outre, permettre aux titulaires d'un contrat à durée déterminée de se maintenir en France pendant au moins un an après l'expiration de leur contrat et d'accéder à la carte de séjour pluriannuelle, comme le suggère l'étude d'impact, pourrait compliquer encore davantage les procédures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière. À la place,

Cette distinction, issue de la loi relative au droit des étrangers de mars 2016, a constitué un recul pour les détenteurs de CDD d'une durée égale ou supérieure à douze mois, puisqu'ils ne relèvent plus de la carte de séjour portant la mention Le monde du travail étant marqué par un recours accru aux CDD, notamment dans les métiers peu qualifiés qu'exercent un certain nombre de personnes étrangères en situation régulière, cette disposition a eu pour effet d'accroître le nombre de cartes de séjour « travailleur temporaire » au détriment des cartes de Or cela constitue un recul pour les travailleurs étrangers, déjà largement précaires, car les droits attachés à l'une et à l'autre cartes ne sont pas identiques. Nous proposons donc de revenir sur cette disposition.

les titulaires d'un contrat à durée déterminée ont une carte de séjour « travailleur temporaire » d'une durée d'un an, puis une carte de séjour pluriannuelle pour la durée de leur contrat. De façon distincte, les titulaires d'un contrat à durée indéterminée

France. Il ne règle en rien la situation de coexistence de deux cartes de séjour concernant des publics très proches, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une complexité assez grande. Comme le Sénat a refusé

Le Gouvernement est défavorable à ces amendements, qui visent à rendre automatique le retrait ou le refus de délivrance d'un titre de séjour en cas de menace pour l'ordre public. En effet, le CESEDA laisse un pouvoir d'appréciation au préfet, lui permettant éventuellement de différer la mesure. Je dois rappeler qu'il est constant que ce dernier retire sans faillir, et dès que possible, le titre de séjour de l'étranger

une capacité d'appréciation. L'an dernier, 197 étrangers en situation irrégulière et 80 étrangers en situation régulière ont fait l'objet d'une mesure administrative d'expulsion.

ces amendements est de prévoir le refus ou le retrait du titre de séjour pour les personnes inscrites au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, le FSPRT. Or, on l'a rappelé, ce fichier est constitué à partir de signalements de concitoyens, voire de simples soupçons, communiqués la ligne téléphonique mise à disposition par le Gouvernement. L'inscription d'une personne dans ce fichier ne fait pas l'objet de vérifications en amont de la part de nos services de renseignement. Il nous manque donc un outil pour retirer directement le titre de séjour des étrangers dont il est prouvé qu'ils sont radicalisés.

Madame la ministre,

prévu par le code des relations entre le public et l'administration. Elle permet ainsi à l'étranger de justifier par écrit ou oralement son absence à la convocation adressée par le préfet, ce dernier ayant la charge d'apprécier le motif invoqué. Votre amendement est donc en fait

Les auteurs du présent amendement ne voient pas où se trouve la simplification avancée par le Gouvernement. Ces exigences supplémentaires leur paraissent, au contraire, alourdir inutilement le CESEDA. Plus grave encore, il semble qu'il s'agisse tout simplement d'une restriction injustifiée du droit au séjour.

Cet amendement vise à préciser la rédaction de l'article 28, qui fixe les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». L'article prévoit que l'étranger doit apporter la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel. Cet amendement vise à poser pour principe que l'étranger dont le montant des ressources est au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel sera présumé pouvoir vivre de ses ressources et n'aura pas à en apporter une preuve. C'est

Ces cartes sont délivrées aux ressortissants étrangers qui viennent en France effectuer une mission dans le cadre d'un détachement afin de suivre un stage, d'occuper un poste d'encadrement supérieur ou d'expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui les emploie. Le salarié conserve son contrat de travail dans l'entreprise du groupe située à l'étranger qui le détache en France. Ces cartes seront désormais non renouvelables et accordées aux seuls étrangers résidant en dehors de l'Union européenne. La durée minimale d'expérience professionnelle au sein du groupe qui emploie le stagiaire est portée à six mois, au lieu de trois actuellement. Un délai de six mois entre la fin d'un transfert temporaire intragroupe en France et une nouvelle demande sera exigé. Le caractère conforme aux prescriptions de la directive du 15 mai 2014 de ces modifications en soi une justification de ce durcissement qui, à l'évidence, ne va pas dans le sens du renforcement de l'attractivité de la France. L'étude d'impact ne donne aucun élément solide justifiant la modification d'un dispositif qui a à peine deux ans d'existence. Elle se limite à évoquer « des suspicions de détournements signalées en 2017 par quelques consulats

Cette mobilité est précisément encadrée par une directive du 15 mai 2014. L'article 29 vient préciser cette transposition en posant un certain nombre

À l'heure actuelle, s'agissant de la disposition visée par la présente modification législative, le 6° de l'article L. 313-11 6° du CESEDA prévoit

qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans L'application de cette disposition se heurte cependant à une suspicion quasiment systématique des administrations préfectorales, eu égard au risque de fraude à la reconnaissance de paternité. Si l'objectif de lutte contre la fraude paraît légitime, le I

en imposant au parent français ayant reconnu l'enfant de démontrer qu'il contribue de manière effective à l'entretien et à l'éducation de celui-ci. Or, une telle mesure risque de porter atteinte atteinte au respect de la vie privée et familiale des personnes étrangères concernées et de constituer une violation du principe de non-discrimination en lien avec la nationalité. De plus, le II de l'article 30 prévoit d'insérer dans le CESEDA cinq nouveaux articles qui créeraient un dispositif d'alerte du procureur de la République par l'officier de l'état civil, à l'instar de ce qui existe pour les suspicions de mariages blancs. L'officier de l'état civil serait ainsi en mesure de saisir le procureur de la République s'il existe des indices sérieux laissant présumer, au vu de l'audition de l'auteur de la reconnaissance de l'enfant, que celle-ci est frauduleuse. Néanmoins, l'absence de définition précise de la notion d'« indices sérieux laissant présumer du caractère frauduleux de la reconnaissance » est problématique, puisque ce dispositif pourrait créer des atteintes non négligeables aux droits des parents et enfants concernés. L'encadrement de cette notion permettrait d'éviter l'automaticité des signalements au parquet, notamment dans l'hypothèse où l'un des parents serait dépourvu de titre de séjour, cette circonstance étant susceptible d'induire une présomption de fraude à l'encontre des étrangers en situation irrégulière. Ces dispositions semblent, en outre, ne pas être nécessaires au regard de l'objectif de lutte contre la fraude, contre la fraude, puisque les dispositifs légaux actuels permettent déjà de faire obstacle aux situations de fraude par l'annulation des reconnaissances frauduleuses, le retrait des titres d'identité ou de séjour indûment délivrés et le recouvrement des prestations indues.

En instaurant une suspicion à l'égard des couples franco-étrangers, le Gouvernement va, en fait, précariser de nombreuses familles et, par ce biais, nombre de femmes et d'enfants. Les auteurs du présent amendement demandent la suppression de l'article 30. La parole

d'une décision du Conseil d'État de 2013, peut tout à fait refuser l'établissement d'un titre de séjour. Nous n'avons donc absolument pas besoin, pour traiter les 3 % de fraudes supposées,

Pour la défense des droits de l'enfant, il est important d'adopter ces amendements.

Il est obligatoire, pour le ressortissant français, de contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant reconnu. Cela ne paraît pas aberrant. En revanche, comme l'a souligné l'Union syndicale des magistrats, la notion de reconnaissance frauduleuse mentionnée au II du présent article n'est définie nulle part, ce qui pourrait rendre délicate l'application de ces dispositions. C'est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer cet article, dans l'attente d'un débat plus approfondi et d'une rédaction plus aboutie.

dans les cas les plus spécifiques, même en l'absence de preuves quant à la contribution effective du père à l'éducation de l'enfant. Cette clause pourrait notamment s'appliquer aux victimes de violences conjugales. Pour ces raisons, j'émets un avis défavorable sur ces trois amendements identiques. Quel est l'avis du Gouvernement ?

de la fraude, il paraît légitime d'exiger une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par l'auteur de la reconnaissance de filiation, ce qui est d'ailleurs conforme à l'intérêt de l'enfant et est exigé de tout parent en vertu des dispositions de l'article 371-2 du code civil. La preuve peut se faire par tous moyens et à proportion des ressources de l'auteur de la reconnaissance de filiation : achats, factures diverses, visites, accompagnement scolaire, etc. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Cet amendement vise à remédier à la situation inadmissible des étrangers qui, bien que résidant en France depuis plusieurs années, sont contraints de vivre en situation irrégulière alors même qu'ils ne peuvent être éloignés du territoire.

parce que ce dernier les refuse. Il faut sortir de cette situation totalement kafkaïenne. Ces personnes se trouvent dans des conditions d'extrême dénuement. Elles vivent à la rue, à l'hôtel ou dans des centres d'hébergement, et ne peuvent accéder à l'emploi ou au logement.

pour essayer de mettre de l'ordre dans les politiques migratoires seraient rendus vains du Gouvernement ? Le préfet dispose d'un pouvoir de régularisation, dont la procédure a été formalisée dans le CESEDA. L'admission exceptionnelle au séjour répond à des conditions fixées fixées par la jurisprudence, au demeurant rappelées au préfet. L'un des critères essentiels est la durée de la présence sur le territoire, sachant que la décision doit se fonder sur un examen global de la situation de l'étranger. Ainsi, l'admission exceptionnelle au séjour permet de prendre en compte la situation de personnes ne remplissant pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sans être pour autant expulsables.

en particulier en Île-de-France, sont aujourd'hui confrontés à des mariages dits « blancs », liés à l'absence de titre de séjour pour l'un des deux mariés. Afin de lutter plus efficacement contre l'immigration irrégulière et, plus particulièrement, contre les mariages blancs, les auteurs de cet amendement souhaitent obliger les élus à signaler au procureur de la République

de la commission ? Le code civil comporte un dispositif de lutte contre les mariages frauduleux : en cas d'indices sérieux, l'officier de l'état civil peut saisir le procureur de la République, qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour se prononcer, délai auquel s'ajoute éventuellement une période de sursis. Le procureur peut s'opposer au mariage, et les intéressés peuvent bien sûr former un recours devant le tribunal de grande instance.

Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition par l'officier de l'état civil de l'auteur de la reconnaissance de l'enfant, que celle-ci est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République et en informe l'auteur de la reconnaissance. » C'est exactement le dispositif que nous souhaitons instaurer pour les mariages qualifiés de « blancs

de la procédure dite des « étrangers malades ». Ce dispositif pourrait se révéler inopérant, l'étranger concerné pouvant s'opposer à un tel échange d'informations entre médecins.

Dès lors, cet amendement tend à autoriser l'échange d'informations entre les médecins traitants et ceux de l'OFII même lorsque l'étranger s'y oppose. En ce sens, nous suivons la logique de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique,

d'assurer l'équilibre du dispositif, les modalités concrètes d'application de ce dernier seraient définies par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la

intéressée. De même, le droit en vigueur prévoit déjà des cas où l'accord des personnes concernées par un échange d'informations n'est pas requis, notamment pour la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail. La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

amendement tend donc à garantir de façon effective que l'autorité administrative ne pourra pas aller contre l'avis du collège de médecins. Hors les cas de menace à l'ordre public ou de fraude, l'autorité administrative sera tenue de suivre l'avis médical : hors ces deux cas, il ne relève pas de la compétence de l'autorité administrative d'apprécier les considérations

qui retarde de façon tout à fait excessive la délivrance de la carte de résident permanent, en prévoyant qu'elle ne peut être délivrée de plein droit qu'à l'occasion du second renouvellement de la carte de résident, soit après vingt-cinq ans de présence régulière sur le territoire français.

permanent, d'une durée indéterminée, qui peut être octroyée à l'expiration d'une première carte de résident. Il s'agit là d'une faculté, et non d'une obligation. En 2016, le législateur a étendu le périmètre de la carte de résident permanent. Désormais, cette dernière est obligatoirement délivrée dès le second renouvellement de la carte de résident simple.

à Mme Claudine Lepage. Cet amendement vise à accélérer le processus de délivrance d'un titre de séjour pour les étrangers victimes de violences conjugales, en supprimant la condition de caractère définitif de la condamnation de l'auteur des faits. Cette condition impose aux victimes de violences conjugales d'attendre que la condamnation soit devenue définitive pour pouvoir prétendre à la délivrance d'une carte de résident.

temporaire. Il n'est donc pas sans titre de séjour. Le Gouvernement ne souhaite pas qu'une carte de résident soit octroyée sans garantie de condamnation pénale définitive de l'auteur des faits,

Cet amendement vise à supprimer la restriction de l'octroi d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » aux seuls bénéficiaires ou anciens bénéficiaires d'une ordonnance de protection.

proposent d'aller encore plus loin : la personne n'aurait plus à demander une ordonnance de protection, le dépôt d'une plainte suffirait. En fait, il convient d'inciter les victimes à solliciter une ordonnance de protection. En effet, cette dernière est bien plus protectrice qu'une simple plainte : elle empêche par exemple tout contact entre la victime et le conjoint violent. Nous craignons que

indéniables, notamment en termes de sécurisation du droit au séjour des victimes de violences conjugales ou d'un mariage forcé bénéficiant d'une ordonnance de protection et des victimes de proxénétisme.

Estimant que la délivrance d'une carte de résident à une personne victime de violences sexuelles ne doit pas être conditionnée au caractère définitif de la condamnation de l'agresseur, les auteurs du présent amendement demandent la suppression de la mention dudit caractère dans la rédaction de l'article. De cette manière, un éventuel appel ne suspendrait pas l'octroi l'octroi de la carte de résident. Il s'agit là d'une condition de la sécurisation effective des exilés victimes de violences sexuelles que le Gouvernement prétend assurer. L'amendement

projet de loi modifie les conditions de délivrance d'une carte de résident pour les étrangers victimes de violences conjugales. Est ainsi prévu l'octroi d'une carte de résident aux seuls étrangers ayant obtenu une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 316-3 du CESEDA. de cette carte de séjour est soumise à l'obtention d'une ordonnance de protection, qui n'est délivrée que trop rarement. Cet amendement vise donc à supprimer cette condition nouvelle, qui prive les victimes de violences conjugales du bénéfice de la carte de résident au seul prétexte qu'elles bénéficiaient jusqu'alors d'un autre titre de séjour que celui qui est prévu à l'article L. 316-3, que ce soit une carte de séjour temporaire portant une autre mention ou une carte de séjour pluriannuelle.

à la condamnation définitive de l'auteur des faits, et de la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'octroi d'une carte de résident. C'est pourquoi le Gouvernement ne souhaite pas que des cartes de résident soient délivrées en dehors de ce nouveau

Cet amendement a pour objet de permettre la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l'étranger qui dépose plainte contre une personne pour des faits de trafic de stupéfiants, de trafic d'armes, de réduction en esclavage ou d'exploitation de la mendicité. Actuellement, l'article L. 316-1 du CESEDA prévoit la délivrance de la carte de séjour portant la

d'un petit système juridique qui, noyé dans le brouillard épais de la suspicion et des, met en cause la protection des femmes de nationalité étrangère dès lors qu'elles auraient l'étrange idée de se séparer de leur conjoint ... C'est là, nous semble-t-il, oublier un peu vite que les discordes familiales ou conjugales n'ont pas de frontières

rectifié. Dans des situations de violences conjugales ou familiales, il importe que l'étranger détenteur d'un titre de séjour en tant que conjoint de Français ou l'étranger admis au séjour dans le cadre du regroupement familial puissent conserver leur droit au séjour s'ils rompent la vie commune pour quitter le contexte familial dans lequel s'exercent des violences. Actuellement, une telle protection de l'étranger victime est prévue en cas de violences conjugales, mais elle ne s'étend pas toujours aux violences familiales ; par ailleurs, elle n'est pas totalement harmonisée entre les conjoints de Français et les conjoints d'étranger entrés en France par le Or la situation de dépendance par rapport au conjoint grâce auquel l'étranger détient son titre de séjour est identique, que les violences soient de nature conjugale ou familiale. En outre, les conjoints de Français et les conjoints d'étranger entrés en France par regroupement familial se trouvent dans des situations identiques, la pérennité de leur titre dépendant dans les deux cas de la communauté de vie avec leur conjoint.

Je rappelle du reste que l'article 33 reprenait des modifications déjà prévues à l'article 203 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, dispositions qui avaient été déclarées inconstitutionnelles, car qualifiées de « cavalier Votre commission des lois a supprimé cet article 33, ce que nous regrettons. Le Gouvernement est attaché au rétablissement de cette avancée en faveur des victimes de violences familiales. La lutte contre les violences faites aux femmes constitue un pilier de l'égalité

objet de supprimer la disposition qui crée, par exception, un titre pluriannuel d'une durée de deux ans pour les étrangers mariés à un ressortissant français, les père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et les étrangers dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser leur séjour porterait à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. La durée dérogatoire prévue n'a aucune justification et a pour effet de maintenir ces personnes dans la précarité, au rebours de l'objectif d'intégration affiché par le Gouvernement.

». Le mécanisme prévu par le texte va à l'encontre de la logique de progressivité du parcours migratoire, en instaurant un va-et-vient entre carte pluriannuelle et carte de séjour temporaire. Cette mesure ne tient pas compte de l'intégration résultant des années passées en France au préalable et enferme les étrangers dans des catégories rigides de droit au séjour.

La loi relative au droit des étrangers en France dispose que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » ou « entrepreneur-profession libérale et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée à un autre titre bénéficie d'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « entrepreneur-profession libérale » lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. L'objectif est de s'assurer que la demande de l'étranger s'inscrive bien dans le cadre d'une démarche professionnelle sérieuse et pérenne. À l'expiration de cette carte de séjour temporaire, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » peut être délivrée à l'étranger s'il remplit les conditions requises. Cependant, s'il satisfait aux conditions de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant en qualité de salarié ou de créateur d'entreprise, cette disposition ne lui est pas applicable ; il pourra bénéficier de cette carte de séjour « passeport talent ». Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable

est une matière relevant de la police administrative. À ce titre, un contrôle important doit être effectué sur les conditions à remplir par l'étranger souhaitant séjourner et, souvent, s'établir sur notre territoire.

lier la possession d'un titre de séjour, dans certains cas précis, au maintien d'une relation conjugale qui peut s'avérer particulièrement difficile, c'est nier l'identité de celle qui en souffre directement et peut fort bien en porter les traces, tant physiquement, quand les violences sont manifestes et corporelles, que mentalement, quand s'y ajoute le mépris découlant d'une relation mal construite, parfois imposée. Soyons clairs pouvons-nous accepter, mes chers collègues, dans la France du XXIsiècle, que la dissolution d'un mariage au mieux arrangé, au pire forcé, ne soit pas un fait justifiant qu'une femme de nationalité étrangère obtienne la protection de la loi, nonobstant le statut finalement accordé ? Les femmes d'origine étrangère qui vivent dans notre pays exercent d'ores et déjà, pour un grand nombre d'entre elles, des activités professionnelles, sociales, économiques, qui leur donnent toute leur place dans la société française. Elles sont, par exemple,

violences. Renouveler le droit au séjour tant que le mariage n'est pas dissous, sans que la rupture de la vie commune puisse être opposée, empêcherait le préfet de sanctionner les mariages blancs ou insincères et favoriserait la fraude. De même, la seule circonstance que le divorce ait été prononcé aux torts du conjoint français ne peut suffire à donner un droit au renouvellement du titre de séjour. Par ailleurs, la communauté de vie en France avec un étranger ou un Français hors mariage n'est pas une condition nécessaire ni suffisante pour obtenir un titre de séjour au vu des liens personnels et familiaux établis en France. L'admission au séjour des ressortissants étrangers victimes de violences de la part de leur partenaire, conjoint ou concubin, est en outre déjà prévue par les dispositions de l'article L. 316-3

pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'État ou des autres collectivités publiques. Cette proposition est issue, en particulier, du rapport du député Aurélien Taché, qui préconise qui préconise de supprimer la condition de nationalité pour l'accès aux concours ouvrant aux fonctions non régaliennes de la fonction publique. C'est aussi une préconisation du Défenseur des droits.

L'abrogation de cette circulaire s'inscrit dans une logique de précarisation accrue de toute une partie de la population parfaitement intégrée, qui étudie, travaille, paye ses impôts, cotise, mène une vie familiale, associative, et qui a vocation à rester sur notre territoire, pour de nombreuses raisons valables et légitimes.

qui régularise une situation irrégulière en raison de sa persistance dans le temps doit être exceptionnelle, et donc rester à la main du pouvoir réglementaire, c'est-à-dire de l'autorité administrative. le pouvoir de régularisation appartient au préfet, qui maîtrise cette procédure. Afin de renforcer la transparence des procédures d'admission exceptionnelle au séjour en clarifiant les éléments d'appréciation des demandes et en favorisant l'harmonisation de leur traitement par les préfectures, la circulaire du 28 novembre 2012, dite circulaire Valls, est venue préciser les orientations générales en matière de régularisation des étrangers, notamment

L'appréciation du préfet doit se fonder nécessairement sur un faisceau d'éléments, l'ancienneté de séjour étant un critère parmi d'autres. Ainsi, le Gouvernement estime que l'article adopté par la commission des lois du Sénat n'apporte en réalité rien sur le plan juridique. En outre, sa rédaction est inopportune, car il ne paraît pas souhaitable de formuler de manière rigide des critères d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour dans une disposition législative.

À partir du moment où l'on admet le droit au séjour d'un étranger en situation irrégulière remplissant telle ou telle condition, on lui donne le droit de se déplacer à l'intérieur de l'ensemble de l'espace Schengen.

qu'une résidence depuis au moins cinq ans sur le territoire français ne saurait justifier à elle seule une admission exceptionnelle au séjour. Certes, les préfets ont une marge de manoeuvre,

La circulaire permet dans une certaine mesure de remédier au caractère arbitraire des décisions. Ainsi, notre amendement tend à étendre son dispositif aux parents dont les enfants sont scolarisés en France, aux personnes justifiant d'un contrat de travail et aux étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur. comme pour les parents d'enfants scolarisés, il s'agit d'une sécurisation et d'une stabilisation importantes, permettant d'envisager une poursuite d'études souple. Il est en effet difficile d'anticiper et de planifier sereinement l'avenir si l'on risque de se voir signifier une obligation de quitter le territoire

conformément à l'article L. 313-14 du CESEDA, du fait de l'évolution très rapide de la situation des personnes concernées. Quel est l'avis de la commission ? L'avis est favorable. Il s'agit de mieux maîtriser les procédures de régularisation.

Une telle évaluation pourrait permettre d'apprécier l'opportunité d'inscrire dans la loi les motifs justifiant une régularisation, afin de passer d'un système de décision discrétionnaire à la consécration

Ainsi, un étranger qui contribue, depuis plusieurs années et de manière réelle et sérieuse, à l'activité d'économie solidaire des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et qui présente des perspectives d'intégration réelles, peut valablement solliciter et, sous réserve qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, obtenir un titre de séjour dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour. En revanche, inscrire explicitement dans la loi qu'un tel motif d'admission au séjour est prévu pour toute personne « présente » dans ces structures

et sans que le préfet puisse s'y opposer, de façon d'ailleurs contradictoire avec les principes mêmes de l'admission exceptionnelle au séjour, qui réservent au préfet un large pouvoir d'appréciation et d'examen des situations dans leur ensemble.

notamment par des filières d'immigration irrégulière. Il convient donc de laisser les préfets user de l'entièreté de leur pouvoir d'appréciation, de sorte que puissent être réglées les situations individuelles signalées par ces associations dans le cadre d'un dialogue avec les préfectures, qui existe dans la plupart des départements et qui permet d'apporter une réponse sociale appropriée à de nombreuses situations, tout en maîtrisant le nombre de régularisations dans leur ensemble.

L'Assemblée nationale a ajouté un dispositif de régularisation d'office pour toutes les personnes qui auraient été accueillies pendant une certaine durée dans une association d'action sociale.

à prévoir un cas de régularisation supplémentaire à l'article L. 313-14 du CESEDA, sur proposition de l'association gestionnaire de l'action sociale, mais sur décision du préfet.

En cas de refus du maire d'inscrire un enfant à l'école -ce sont des choses qui arrivent -, le code général des collectivités territoriales prévoit que le préfet procède lui-même à l'inscription ou enjoigne au maire de le faire. Une telle intervention du préfet n'est cependant possible que s'il est informé du refus d'inscrire l'enfant. Or, pour les familles néo-arrivantes- mais pas uniquement elles -, il peut être difficile de connaître les démarches administratives à effectuer pour faire valoir le droit à l'éducation Il est donc important de prévoir un dispositif d'urgence en pareil cas, visant à assurer que la scolarisation de l'enfant soit effective. Cet amendement tend donc à rétablir la disposition adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale et à imposer que, en cas de refus du maire, celui-ci en informe immédiatement le directeur académique des services de l'éducation nationale, qui autorisera l'accueil provisoire de l'enfant et sollicitera le préfet pour procéder à une inscription définitive.

Le refus de scolariser les enfants étrangers sur des fondements illégaux est d'ailleurs déjà sanctionné par les tribunaux administratifs, qui peuvent enjoindre aux maires, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder aux inscriptions. Il n'y a donc pas lieu de prévoir de procédure d'urgence supplémentaire. En revanche, il appartient en effet au préfet et aux services de mettre en oeuvre les prérogatives qu'ils tirent de la loi et de prêter toute l'attention nécessaire aux cas d'espèce,

de finances. Étonnamment, contrairement aux conjoints extracommunautaires de ressortissants de l'Union résidant en France, les conjoints étrangers de Français qui souhaitent obtenir une première carte de séjour ont l'obligation de produire un visa de long séjour.

Or, lorsqu'ils sont contraints de retourner dans leur pays d'origine, les conjoints de Français qui sont dans ce cas doivent souvent patienter plusieurs mois avant d'obtenir leur visa. J'ajoute que le dispositif actuel a pour effet de contraindre des conjoints à vivre séparément, parfois pendant de longues périodes, ce qui n'est pas souhaitable. qui n'est pas souhaitable. De ce fait, il contribue à fragiliser le droit de mener une vie familiale normale, qui repose, comme le stipule la Convention européenne des droits de l'homme, sur la vie en commun.

à M. Xavier Iacovelli. Actuellement, l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit trois conditions cumulatives pour l'obtention d'un visa de long séjour sur place pour les étrangers mariés à des ressortissants français

ou ne peuvent pas justifier d'une entrée régulière, ils ne peuvent obtenir le visa de long séjour sur place et doivent retourner dans leur pays d'origine pour cela. Certaines personnes sont cependant dans l'impossibilité de retourner dans leur pays d'origine et sont donc maintenues en situation irrégulière en France, sans pouvoir être expulsables car elles sont les conjoints de ressortissants français.

inextricable de ces personnes qui ne sont ni régularisables ni expulsables.

ne peuvent pas déposer leur demande de visa de long séjour auprès de la préfecture, y compris lorsque le mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français. Cela signifie par exemple qu'une ressortissante argentine ayant épousé un Français au Mexique au Mexique est contrainte, pour pouvoir résider sur notre territoire avec son conjoint, de repartir à Buenos Aires afin d'y solliciter la délivrance d'un visa de long séjour auprès du consulat. L'obligation de détenir un visa de long séjour est préjudiciable à la vie des couples binationaux. Elle a notamment pour effet de priver les enfants d'un de leurs parents pendant une période qui peut être assez longue. Cette situation n'est pas acceptable au regard du droit à mener une vie familiale normale. Je vous propose, mes chers collègues, de mettre un terme à cette différence de traitement en adoptant le présent amendement.

de Français. Ce sujet est important puisque, chaque année, environ 40 000 conjoints de Français sont admis au séjour. Il s'agit du premier motif d'immigration familiale. L'amendement n° 174 rectifié tend à supprimer l'obligation, pour le conjoint de Français, de produire un visa afin d'entrer en France. Certes, lorsque l'étranger est marié à un Européen, son conjoint n'a pas à produire de visa, mais cette dérogation est justifiée par le fait qu'il est européen, non par celui d'être le conjoint d'un Français. En outre, depuis 2006, un conjoint de Français peut solliciter un visa à la préfecture sans retourner dans son pays d'origine, à trois conditions : il est entré régulièrement en France ; le mariage a été célébré en France ; il vit en France depuis plus de six mois avec son conjoint.

L'instruction d'une demande de visa de long séjour n'a pas pour effet de rendre l'accès au séjour des conjoints de Français plus Pour l'obtention d'un tel visa, le demandeur doit justifier de sa situation matrimoniale, ainsi que de la nationalité française de son conjoint. Un refus de visa ne peut être opposé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. La suppression du visa de long séjour pour les conjoints de Français aurait pour effet de rendre inopérantes les procédures de contrôle préalables à toute entrée sur le territoire français, sachant que les conjoints de Français représentent la première catégorie

vise à rétablir le dispositif accordant le bénéfice de l'extension de validité de trois mois dans l'attente du renouvellement d'une carte aux titulaires d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximum de quatre ans, d'une part, et aux titulaires d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée inférieure à quatre ans, Le rapporteur a supprimé ce dispositif au motif que son impact n'était pas suffisamment évalué. Or cette évaluation a vocation à s'opérer progressivement à l'occasion de l'expérimentation prévue pour trois ans dans un nombre limité de départements, dont la liste serait définie

À l'expiration de sa carte de résident d'une durée de dix ans, un étranger peut justifier de la régularité de son séjour pendant un délai de trois mois, notamment pour éviter des « ruptures de droit pour objet d'étendre ce dispositif aux cartes de séjour pluriannuelles et aux cartes de séjour temporaires. Or, cette mesure emporterait un certain nombre d'effets non désirés. À titre d'exemple,

Il prévoit également la possibilité d'un retrait du titre en cas de retrait du certificat de bonne conduite, par exemple pour cause de désertion. Il s'agit de tenir compte de l'engagement singulier de la Légion étrangère au service de la France, hier et aujourd'hui. Tous ses membres servent en opérations extérieures au cours de leurs cinq premières années d'engagement. Par ailleurs, cet amendement prévoit un mécanisme destiné à éviter que l'attribution facilitée d'un titre de séjour ne conduise à créer une nouvelle voie d'immigration, en s'assurant que la personne concernée continue bien à exercer ses fonctions au sein de la Légion.

C'est un amendement de coordination, monsieur le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

entre le territoire métropolitain et les territoires ultramarins, notamment Mayotte, où les dispositions dérogatoires au droit commun sont les plus choquantes. Nous avons bien conscience, compte tenu des amendements visant à adapter le droit

En outre, les zones d'attente à Mayotte peuvent être des zones de prison, relevant donc de l'administration pénitentiaire. Enfin, l'existence d'une commission du titre de séjour en Guyane, à Mayotte et à Saint-Martin pose question. Comment l'expliquer, si ce n'est par le désintérêt, voire le mépris, pour les demandes des ressortissants étrangers, qui méritent pourtant un examen exhaustif ? En parallèle, il devrait être procédé à l'abrogation de dispositions réglementaires qui instaurent une inégalité de traitement inacceptable entre étrangers selon le lieu du territoire de la République où ils se trouvent. Si nous comprenons que certaines que certaines adaptations peuvent théoriquement être rendues nécessaires au regard des spécificités ultramarines, nous n'acceptons pas ces différences de traitement qui rompent l'égalité entre les citoyens.

Gouvernement ? Même avis. Les articles du CESEDA visant à prendre en compte les spécificités de Mayotte sont utiles. En effet, l'écart de conditions de vie entre Mayotte et son environnement régional est à l'origine d'une forte pression migratoire sur ce département, et des mesures d'éloignement spécifiques sont donc nécessaires compte tenu du nombre important d'étrangers en situation irrégulière. En outre, la jurisprudence administrative a confirmé que le dispositif actuel ne contrevient ni au principe d'égalité et d'indivisibilité de la République ni à la liberté d'aller et de venir. La parole est à

Il est impossible de définir une solution uniforme applicable aux situations extrêmement différentes que nous rencontrons de Calais à Menton, en passant par Paris, la Guyane et Mayotte.

insérée dans un bassin géographique sud-américain marqué tant par l'instabilité politique que par les difficultés économiques et environnementales, il est rarement question de victimes de guerre ou de réfugiés politiques, mais plutôt de femmes et d'hommes venus chercher une vie meilleure.

s'agissant du droit d'asile à proprement parler, comment ne pas considérer qu'il est aujourd'hui dévoyé en Guyane, littéralement pris en otage par des filières d'immigration clandestine ? C'est donc le droit à la différenciation que je défends ici, parce que la Guyane et Mayotte se démarquent, chacun à sa manière, du reste du territoire français. L'accélération des délais de traitement doit permettre, d'une part, de mieux traiter les demandes légitimes, et, d'autre part, de réduire l'attractivité de ces Enfin, il me semble indispensable d'organiser la coopération sanitaire avec les pays voisins, afin de soulager la pression migratoire qui pèse actuellement sur nos établissements de santé.

Éric Kerrouche. Cet amendement vise à préciser le mode de désignation des trois députés et des trois sénateurs membres de l'Observatoire de l'asile, chargé d'évaluer la politique de l'asile dans les départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Par cet amendement, nous proposons de supprimer la prolongation de la dérogation à l'obligation de séparer les locaux affectés à la rétention administrative et au maintien en zone d'attente à Mayotte. Nous connaissons la situation à Mayotte

Il s'agit de faire preuve de cohérence : soit Mayotte est dans une situation telle que la pression migratoire qu'elle subit n'est plus tolérable, et dans ce cas l'adoption de cet amendement est indispensable soit ce qui se passe à Mayotte n'est pas grave, et je ne vois pas en quoi les dispositions de cet amendement constitueraient une menace pour le reste du territoire et pourquoi elles ne pourraient pas être adoptées.

Il nous semble que vous envisagez le problème à l'envers et que vous cherchez à lisser la situation dans un sens défavorable au département de Mayotte, en restreignant en outre la circulation des mineurs, au lieu d'ouvrir celle des adultes.

de quitter rapidement l'archipel pour rejoindre le continent européen ne ferait que renforcer le caractère attractif de ce département pour les ressortissants des États voisins. Le risque de détournement des procédures

Comment voulez-vous résoudre le problème de la pression migratoire à Mayotte si l'Hexagone n'est pas solidaire ? Or émettre des avis défavorables sur cet amendement, c'est signifier

!On ne peut pas transformer un département français en centre de rétention à ciel ouvert.

est à M. Claude Malhuret. Les migrations ne sont pas évoquées à l'article 1 de la loi d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale, qui définit les objectifs de l'aide au développement française. Cette omission est d'autant moins compréhensible qu'il est avéré que le sous-développement et la pauvreté sont des causes fondamentales des migrations, et que seule une stratégie structurelle, agissant sur la capacité des pays sources à donner un avenir à leur jeunesse, pourra nous permettre de lutter efficacement contre la crise migratoire que nous connaissons. Cet amendement vise donc à préciser explicitement que l'aide au développement française contribue à lutter contre les causes des migrations.

Toutefois, l'article 3 de cette loi prévoit de rechercher une cohérence entre les objectifs de la politique de développement et de solidarité internationale et ceux des autres politiques publiques susceptibles d'avoir un impact dans le domaine migratoire. L'article 2 de cette même loi approuve un rapport annexé fixant les orientations de la politique de développement et de solidarité internationale. Ce rapport comprend un volet intitulé « Mobilité, migrations et développement ».

aux collectivités de Wallis-et-Futuna, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Nous considérons que le Parlement doit être saisi de ces questions qui concernent le code de la nationalité et qu'il ne peut y avoir de transfert de compétences par ordonnance au Gouvernement

en Guyane, compte tenu des caractéristiques et des contraintes particulières de ce territoire, qui entraînent, en matière d'asile, une situation différente de celle des autres collectivités françaises. Je vous rappelle que la Guyane n'est pas dans l'espace Schengen

Parallèlement, le décret n° 2018-385 du 23 mai 2018 portant expérimentation de certaines modalités de traitement des demandes d'asile en Guyane prévoit également de nouvelles mesures dérogatoires au droit commun. L'expérimentation prévoit notamment de réduire à sept jours, au lieu de vingt et un, le délai dans lequel le demandeur d'asile doit déposer sa demande à l'OFPRA,

Pour rappel, en dépit des chiffres précités, la Guyane ne dispose d'aucun centre d'accueil de demandeurs d'asile, ou CADA, et la majeure partie des cent places d'hébergement d'urgence disponibles sont réservées aux familles. Cette faible capacité d'hébergement n'est pas sans conséquence sur la prolifération de l'habitat illicite, qui transforme la périphérie de nos villes en véritables bidonvilles. De même, l'accueil des enfants est source de grandes difficultés dans l'académie de Guyane à chaque rentrée scolaire, le Centre académique d'enfants allophones nouvellement arrivés étant totalement saturé. l'accélération des délais de traitement pose avec acuité la question de l'interprétariat, indispensable pour permettre aux demandeurs d'asile de remettre à temps un dossier complet en langue française. de cet amendement proposent que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de dix-huit mois, un rapport sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Guyane.

En effet, depuis des années, que ce soit dans les accords de Paris ou avec l'initiative Nansen, les changements climatiques sont reconnus comme une menace à l'échelle mondiale, dont les conséquences pesant sur l'humanité se traduiront bientôt par des mouvements intenses de populations aux échelles nationale et internationale. Face à la répétition de ces crises, il est donc urgent de clarifier les motifs conduisant des personnes à demander l'asile sur notre territoire. C'est pourquoi nous proposons de supprimer symboliquement l'article 42 du projet de loi dans sa rédaction actuelle, afin de souligner son

ministre. La répartition des compétences entre la CNDA et les tribunaux administratifs fait l'objet de deux types de critiques. D'une part, la répartition du contentieux des décisions de l'OFPRA du droit d'asile paraît complexe et a suscité des incertitudes de jurisprudence. Si celles-ci sont partiellement levées, il peut être pertinent de s'interroger sur la nécessaire simplification de ce droit. D'autre part, le projet de loi, en permettant au tribunal administratif statuant sur une OQTF de donner, le cas échéant, un effet suspensif au recours devant la CNDA, a introduit une complexité supplémentaire. Il convient toutefois, sur cette matière complexe, de prendre le temps de l'étude et de la concertation, avant de savoir quelle réforme serait appropriée. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a déposé cet amendement, qui vise à

; enfin, à garantir que, quelle que soit la réforme, celle-ci ne visera pas à revenir sur la spécificité de la compétence de la Cour nationale du droit d'asile, dont le modèle doit être préservé. Il s'agit donc d'un amendement visant à aboutir, au terme d'un travail d'étude auquel le Parlement sera associé, à une réforme technique, si celle-ci est nécessaire.

contentieux des décisions de l'OFPRA et du droit de se maintenir sur le territoire. Il propose au même moment de l'habiliter à modifier par voie d'ordonnance les dispositions législatives relatives à ce contentieux dans les deux prochaines années. Le Gouvernement justifie ces mesures introduites devant le Sénat par les critiques dont a pu faire l'objet la répartition de ce contentieux, s'agissant notamment de l'article 8, qui prévoit un mécanisme de contestation de l'OQTF devant le juge administratif, alors que le demandeur a fait un recours non suspensif devant la CNDA. Le procédé utilisé me semble étonnant : on ne peut pas saisir ce prétexte pour dessaisir le Parlement de sa compétence sur la répartition de ce contentieux,

de la recomposition des compétences et, dans le même article, demander, avec beaucoup d'avance et peu d'indications sur le contenu, une habilitation dont l'application se produirait dans un délai compris entre deux ans et deux ans et demi n'est pas la meilleure méthode. Il me semble que le Gouvernement serait mieux inspiré de produire le rapport sur lequel vont travailler les membres du Conseil d'État, les représentants des tribunaux administratifs et les représentants de la CNDA, ainsi, éventuellement, que d'autres experts, puis, sur la base de ce rapport, de nous convaincre

Le Gouvernement a déposé cet amendement à la demande du Conseil d'État. Alain Richard ayant pris la position qu'il a prise, je me sens autorisée à le retirer

Nansen et de l'agenda pour la protection des personnes déplacées en contexte de catastrophes et de changement climatique, adopté à la fin de 2015 par 110 pays, lors des travaux préparatoires à la COP21 et aux accords de Paris. Nous proposons une rédaction simplifiée, qui s'inspire de la définition de l'Office international des migrants. Je la cite : « Les migrants environnementaux sont des personnes ou des groupes qui, pour des raisons de changements soudains ou progressifs de l'environnement qui ont affecté leurs conditions de vie, sont obligés de quitter leur foyer, ou choisissent de le quitter, temporairement ou de manière permanente, et qui se déplacent à l'intérieur des frontières de leur pays ou au-delà. ou au-delà. » Il est proposé de créer un visa temporaire de réfugié climatique à la suite de catastrophes naturelles ou liées à l'activité humaine, avec trois causes limitatives d'accès à ce statut : changement climatique, catastrophe industrielle et catastrophe naturelle.

même pays. Je rappelle que la France est très active à l'échelle internationale sur ce sujet. Par ailleurs, le projet de loi prévoit par ailleurs l'élaboration d'une stratégie nationale de prise en compte des migrations climatiques.

qu'ils soient précis et affichés ! C'est la raison pour laquelle je vous propose l'intitulé de projet de loi suivant : « Projet de loi tendant à renier les engagements de la France en matière d'accueil des réfugiés et à restreindre le droit des étrangers et leur intégration ». Au moins les choses sont claires, et nous faisons ce que nous disons.

Le droit d'asile, que personne dans cette assemblée ne conteste, doit être mis à sa juste place. En aucun cas, il ne doit être le prétexte à une immigration économique et massive, exploitée par des filières de passeurs et par des associations complices. Madame la ministre, j'ai lu attentivement l'exposé des motifs de votre texte. À aucun moment, vous ne faites référence à notre histoire, à notre culture, à notre identité. Pourquoi ? Est-ce une omission volontaire ? Pis, votre projet de loi est agrémenté de mesures permissives, comme l'élargissement du regroupement familial aux frères et soeurs de mineurs réfugiés, dont certaines dispositions ont été corrigées par la commission des lois du Sénat, alors même que de nombreux mineurs étrangers viennent largement alimenter les violences urbaines- quelque 195 000 faits ont été dénombrés en 2017, soit plus de 21 % sur la totalité des infractions constatées. La France doit pouvoir retrouver la maîtrise de son destin en matière d'immigration. Elle doit être libre de choisir qui elle accueille et refuse sur son sol. Elle doit pouvoir faire appliquer ses lois en expulsant les immigrés clandestins. Elle n'est pas un supermarché à prestations sociales. Mes chers collègues, l'objet de cet amendement est de nommer les choses, sans langue de bois. Nous ne devons pas craindre de dire ce que nous voulons combattre- l'immigration massive et clandestine et ce que nous voulons défendre- nos traditions, l'égalité entre les sexes, le respect de la loi, notre belle histoire, notre civilisation, bref, notre identité française. Inscrivons

Je crois avoir compris, au travers des propos de certains, que les immigrés

chers collègues, étaient naturellement réparties sur le globe à l'origine. Des conquérants cupides ont tout déréglé en évitant de rencontrer l'autre, mais en prétendant l'avoir découvert, non sans s'être posé la question de son rang dans une hiérarchie des humanités, dont ils ont vite fait de prétendre être le sommet. La suite, triangulaire, nous a très rapidement renseignés sur la réponse ... Les immigrants ne font que suivre leurs richesses pillées, emportées et transférées.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, devant tant d'aveuglement et de discours sur l'histoire longue, je vous invite à nous pencher sur notre histoire, l'histoire de la France. Comment ne pas penser en ce moment à Michel Poniatowski ?

-que Mayotte et la Guyane aient des dérogations. Eh bien, ce que je demande pour Mayotte et la Guyane, je le demande aussi pour l'ensemble de la France ! Aujourd'hui, nous savons tous que nous sommes menacés par une partie de la population que nous laissons s'installer

Cette âme, la France est en train de la perdre, non seulement à cause de la mondialisation, mais aussi, et surtout, à cause de la société à la fois pluriethnique et pluriculturelle que l'on s'acharne au nom de fausses idées et de vrais mensonges à lui imposer.